Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Mon groupe a inscrit dans son espace réservé de cet après-midi une proposition de loi, adoptée le 2 février 2017 à l'Assemblée nationale, qui permet une revalorisation sensible des retraites agricoles. Cette proposition de loi est attendue par le monde rural tant est grand le dénuement des agriculteurs après une vie passée au service de notre pays et de nos territoires- car que serait la France sans leur travail ? Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité en commission des affaires sociales. Son adoption conforme et donc définitive était acquise. C'était sans compter l'obstination antisociale du Gouvernement, qui, ce matin et ce matin seulement, a déposé un amendement en annonçant un vote bloqué sur ce texte, dans le cadre de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution. En clair, le coup de force du Gouvernement est de n'autoriser l'adoption de ce texte qu'accompagné de l'amendement proposé. Or cet amendement, c'est l'enterrement du texte, puisqu'il reporte son application, voire son existence même : le Gouvernement entend vérifier la compatibilité de la proposition avec la future réforme des retraites De toute façon, la poursuite de la navette n'aura pas lieu, car le texte, qui sera non conforme, ne sera pas inscrit par le Gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Monsieur le président, mes chers collègues, il s'agit d'un coup de force d'une rare violence contre le Parlement ! C'est un coup de force inédit, car l'article 44, alinéa 3,

cela fait des années que nous alertons sur le recul des pouvoirs du Parlement, sur son abaissement. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous parvenons à un moment grave pour notre démocratie, face à la volonté d'Emmanuel Macron d'accaparer tous les pouvoirs. Le Gouvernement doit ! -abandonner le recours au vote bloqué, qui va provoquer l'enterrement de cette proposition de loi. Nous vous demandons de réunir dans l'urgence une conférence des présidents pour permettre au Sénat de riposter dans la plus large unanimité possible face à ce coup de force

Monsieur le président, si je vous ai demandé la parole, ce n'est pas pour vous dire combien il est urgent de revaloriser les retraites agricoles. Je crois que nous partageons ce point de vue sur toutes les travées, tant nos retraités de l'agriculture ont aujourd'hui des revenus qui les pénalisent par rapport aux autres Français, après une vie de labeur souvent commencée, sans qu'elle puisse être prise en compte, avant l'âge de seize ans. Si je prends la parole, c'est parce que, dans notre Haute Assemblée, la commission des lois est aussi celle du Règlement, avec un R majuscule, qui désigne le règlement du Sénat. Je voudrais m'associer à ce rappel au règlement et des comptes publics, que je n'ai pas connaissance de précédents de l'utilisation de cet article 44, troisième alinéa, relatif au vote bloqué depuis de très nombreuses années, et jamais autrement que pour faire aboutir un projet du Gouvernement lorsque la discussion est difficile. L'opposer aujourd'hui à la discussion d'une proposition de loi d'origine parlementaire adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale constitue, de mon point de vue, un précédent extrêmement

en prenant cette décision, que je crois être largement improvisée. Très bien ! C'est la raison pour laquelle je vous demande à mon tour, solennellement, de prendre dans la journée la décision nécessaire pour que le débat ait lieu et qu'il puisse aboutir. Car c'est mal augurer de l'avenir de nos discussions sur le travail législatif que de procéder par l'utilisation de moyens qui exercent sur le Parlement un rapport de force tout à fait inadmissible. Je dois vous dire aussi ma conviction profonde que le recours à ces instruments de rationalisation du parlementarisme, alors qu'il n'y a pas, dans notre pays, de problèmes de majorité pour le gouvernement actuel, est un aveu de faiblesse ! Tout à fait ! Si le Gouvernement avait des arguments pour convaincre le Parlement, il n'aurait pas besoin de recourir à de tels artifices dans la procédure législative. Pardonnez la véhémence et la solennité de mon propos, mais je crois que le sujet est grave. Nous ne pouvons pas laisser passer ce type de décisions unilatérales, non précédées de concertation, et dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel on utilise habituellement- et le moins souvent possible, d'ailleurs -le troisième alinéa de l'article 44 de notre Constitution.

ont été faites hier laissent mal augurer de la suite. Alors qu'une réforme constitutionnelle doit être une réforme apaisée, celle-là s'annonce tout de même bien mal ! On confond vitesse et précipitation ; on confond légiférer vite et légiférer bien

son incompréhension, dans un contexte général de volonté de passer en force et de ne pas mener les débats devant le Parlement.

toute affaire cessante M. le Premier ministre pour l'informer de la situation qui prévaut au Sénat à la suite de ce rappel au règlement. Je souhaite qu'il puisse le faire dès maintenant, car il y a urgence, puisque le texte concerné est inscrit à notre ordre du jour de la fin de l'après-midi.

et républicain, de la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi, présentée par M. Franck Montaugé

les deux textes que j'ai le plaisir de vous présenter cet après-midi au nom de mon groupe répondent à l'objectif, que je crois largement partagé, d'améliorer la qualité de la loi et le suivi de ses effets. L'exécutif, le législatif, les autorités de contrôle et les citoyens sont directement concernés par ce sujet, dans un contexte national et international qui nous amène à penser l'évaluation des normes et des politiques publiques dans le rapport aux enjeux du développement durable

La recommandation centrale de ce rapport, qui a fait date et autorité, est que la croissance est soutenable quand on transmet aux générations futures un patrimoine national susceptible d'assurer la couverture de leurs besoins et de garantir sur le long terme leur bien-être. Cela suppose de pouvoir évaluer le patrimoine national en recensant les divers types de capitaux ou d'actifs qui le composent, en stock et en flux, au nombre desquels figurent le capital économique, privé et public, qui est composé du capital productif ; le capital humain, qui renvoie au niveau d'éducation de la société, aux compétences, au niveau de formation et de qualification du travail ; le capital social, qui est un actif intangible mesurant la qualité des institutions et des rapports sociaux, comme la culture ou le mode d'organisation de la société- il s'agit d'ailleurs d'un indicateur permettant de mesurer le degré de cohésion de la société -et le capital naturel, qui est composé des ressources naturelles, comme les énergies fossiles, l'eau, les terres, et l'ensemble des écosystèmes. Certains économistes ajoutent encore à ce bilan patrimonial de la Nation un actif intangible, comme la démocratie. Au passif du bilan patrimonial de la Nation figurent la dette publique et la dette privée. Pour Jean-Paul Fitoussi, disposer d'un tel bilan patrimonial de la Nation permet d'éclairer les choix politiques, notamment les choix budgétaires. C'est en cela que cette approche nous concerne tout particulièrement. Dans le même esprit, la loi portée par la députée écologiste Éva Sas permet depuis 2015 de « prendre en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques Ce texte a été une première étape importante dans la reconnaissance d'indicateurs permettant de mesurer différents aspects de notre développement : le taux d'emploi, l'effort de recherche, l'endettement, l'espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie, les inégalités de revenus, la pauvreté en conditions de vie, les sorties précoces du système scolaire, l'empreinte carbone et l'artificialisation des sols. Dans l'édito du troisième rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, que nous venons de recevoir,

le Premier ministre : « Cette dynamique [ ...] a un sens politique profond. Il s'agit de savoir ce sur quoi nous fondons collectivement notre appréciation de ce que l'on entend par croissance, développement, bien-être ou progrès. » il indique que les principales réformes engagées par le Gouvernement seront « évaluées à l'aune de ces indicateurs ». Si nous suivons les propos du Premier ministre, l'utilisation des nouveaux indicateurs de richesse de la loi Sas dans les études d'impact, comme le prévoyait notre article 1, n'était pas incongrue. la réintroduction de l'article 1 initial permettrait facilement de surmonter la contradiction entre les propos du Premier ministre et la position de la commission des lois.

Comment nous, parlementaires, pourrions-nous mieux appréhender ces objectifs dans la mise en oeuvre des différentes politiques que nous examinons ? » La nécessité de territorialiser ces indicateurs, d'y associer la société civile, de faire en sorte que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent y travailler ensemble- c'est tout le sens de notre proposition, pour le deuxième texte, d'un Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être -que nos commissions organiques ou spéciales ne travaillent plus en silo était rappelée à juste titre par Jérôme Bignon. En 2011, l'OCDE se dotait d'une démarche du même ordre, intitulée, permettant des comparaisons internationales sur des thèmes aussi importants pour la qualité de vie de chacun de nos concitoyens que l'emploi et les salaires, le rapport vie professionnelle/vie privée, le logement, la qualité de l'environnement, l'état de santé, l'éducation et les compétences, les liens sociaux, l'engagement civique et la gouvernance, la sécurité personnelle et tout ce qui relève du bien-être subjectif. L'Union européenne a aussi développé son propre modèle, et de nombreux pays se sont engagés dans cette voie, chacun à leur manière. En réalité, il y a beaucoup d'indicateurs et de systèmes différents. Cette profusion nuit au sens, à la compréhension et à l'appropriation. Et tant que nous n'avançons pas dans ce sens, le PIB reste le point de repère exclusif, si ce n'est l'objectif majeur. Dans ce contexte, confortés par de nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons ouvert le vaste chantier de l'amélioration de la fabrique de la loi et de l'évaluation des politiques publiques.

« l'ardente obligation de bien suivre l'application des lois en s'assurant de leur pertinence dans la durée, de leurs effets dans le temps pour les corriger ou y revenir ». De son côté, le président du Sénat indique dans la présentation du rapport de François Pillet que le contrôle et l'évaluation ont jusqu'à présent été les « parents pauvres de V République » et que nous devons « davantage investir notre mission de contrôle et d'évaluation ». C'est là tout le sens de nos propositions ! Venons-en maintenant au fond du texte. Dans sa version initiale, l'article 1 de la proposition de loi dont nous allons discuter prévoyait que les études d'impact soient réalisées de manière plus qualitative, en tenant compte des indicateurs de la loi Sas. Nous voulions, à partir de l'usage de ces indicateurs dans les études d'impact, rappeler la nécessité de penser l'action publique au regard des objectifs de développement durable que notre pays reconnaît dans le cadre des accords de Paris issus de la COP 21. Les indicateurs de la loi Sas ne sont pas gravés dans le marbre, mais ils peuvent être mis en rapport avec les dix-sept objectifs de développement durable. Ces « ODD » nécessitent une déclinaison et une appropriation par chaque pays les nouveaux indicateurs de richesse de la loi Sas peuvent en être une traduction pertinente et, bien entendu, perfectible. Ce qui importe donc, pour être cohérents avec nos engagements internationaux, c'est que nous nous engagions à les prendre en compte, à nous y référer dans nos études d'impact et nos évaluations. Là était l'esprit de l'article 1, c'est-à-dire, en réalité, l'essentiel de ce texte. La discussion de l'amendement visant à le réintroduire dans le texte nous permettra, je l'espère, de mieux nous comprendre et d'arriver à un accord. Le rapporteur Le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Jean-Pierre Sueur, a voulu privilégier dans ce texte l'amélioration de la procédure des études d'impact dont traite l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Ce point de vue n'est pas contradictoire avec la réintroduction de l'article 1. -c'est un point important -que « les évaluations sont réalisées par des organismes indépendants ». Nous sommes d'accord avec cette disposition, mais, par cohérence avec la nécessité de faire usage de nouveaux indicateurs, nous amenderons le point relatif aux modalités de réalisation des évaluations.

Nous expliciterons ce point en présentant un amendement de réintroduction de cette notion. La commission des lois a aussi voulu confier au Conseil d'État le soin de définir la liste des organismes habilités, les modalités de leur désignation et les modalités techniques de réalisation des études d'impact et d'évaluation.

Enfin, constatons ensemble que les autres modifications introduites par la commission reposent sur la prise en compte des propositions 15 et 18 du rapport du président Gérard Larcher, relatives à l'amélioration de la qualité des études d'impact. En définitive, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, l'adoption du texte dont la commission s'est saisie ferait, je le crois, progresser sensiblement le Parlement dans la mise en oeuvre des missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques que lui confère l'article 24 de la Constitution, cela dans le cadre d'un paradigme qui répond aux enjeux impérieux d'un développement durable et inclusif. La France a donné la meilleure image d'elle-même avec l'Accord de Paris. Il nous revient, à nous parlementaires, d'en tirer toutes les conséquences dans notre travail quotidien de législateur.

Nous avons également retenu trois amendements émanant du groupe de travail mis en place par le président Larcher et dont François Pillet était le rapporteur : le premier porte sur les moyens mis en oeuvre par le projet de loi,

a instauré le Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités locales, présidé par M. Alain Lambert. Il s'agit d'une instance très utile, car elle permet aux représentants des élus locaux de s'exprimer en amont

Voilà, mes chers collègues, comment, à partir du travail important de Franck Montaugé et de la commission des lois, nous sommes parvenus à un accord sur le texte maintenant soumis à votre approbation. La parole

Ces propositions de loi tendent à améliorer deux phases de la procédure législative : en début de parcours, la présentation des projets de loi par le Gouvernement et la qualité de l'information qu'il produit à l'attention du Parlement au travers des études d'impact ; à l'issue du vote des assemblées, l'évaluation des politiques publiques et de la législation, à l'aune de nouveaux indicateurs de richesse prévus dans la loi dite « Sas » du 13 avril 2015. Le Gouvernement entend saluer, comme l'a d'ailleurs fait la commission des lois, la cohérence et la qualité du travail accompli par l'auteur de ces textes, Franck Montaugé, ainsi que par le groupe socialiste et républicain, qui ont cherché à améliorer l'ensemble du processus législatif, en voulant que le Parlement soit mieux informé, ou informé différemment, à l'occasion du vote des projets de loi qui lui sont soumis, et mieux doté en outils de contrôle de l'application des textes votés et d'évaluation des politiques publiques. C'est la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi que nous allons d'abord examiner. Ce texte est né d'une déception, que le Gouvernement peut entendre. Le parlementaire que j'ai été le sait les études d'impact prévues par le législateur organique dans la loi organique du 15 avril 2009, qui sont censées éclairer le Parlement sur la pertinence du recours à une nouvelle législation, ne sont pas toujours à la hauteur des attentes qui avaient été placées en elles. Perçues à l'origine, lors de la révision constitutionnelle de 2008, comme une clé pour mieux légiférer, elles peuvent parfois apparaître comme incomplètes, biaisées ou, pour le dire autrement, orientées. Je sais que le Sénat est particulièrement vigilant sur ce sujet. Votre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, désormais membre du Conseil constitutionnel, n'a jamais vraiment tenu ces études d'impact en haute estime. Hugues Portelli, éminent professeur de droit public et de sciences politiques, a en outre remis en 2015 sur ce sujet un rapport qui a fait date.

mais il s'agit d'un aiguillon, d'un stimulant indispensable pour améliorer le travail normatif et pour trouver, ensemble, des réponses à une situation perçue comme insatisfaisante. La proposition de loi organique que nous examinons cet après-midi s'inscrit dans la lignée des travaux engagés par le Sénat pour améliorer la qualité des études d'impact. Elle vient s'ajouter à une proposition de loi organique relative aux études d'impact des projets de loi déposée le 28 septembre 2017 par Mme Élisabeth Lamure et M. Olivier Cadic. Son ambition est de permettre une évaluation plus qualitative des projets de loi, par l'intégration dans les études d'impact de nouveaux indicateurs et, pour la réalisation de ces études, par le recours à des organismes indépendants, ainsi qu'à des personnalités qualifiées désignées par le Parlement.

En premier lieu, le Gouvernement ne peut être favorable, par principe, à un texte qui, bien que sensiblement modifié par la commission des lois, ne correspond pas aux orientations données par le Président de la République dans le cadre de la révision constitutionnelle. Sans nier l'intérêt qu'il y a, pour le Parlement, à disposer de la meilleure information possible avant de voter sur un projet de loi, le Gouvernement considère en effet que les dispositions déjà existantes concernant les études d'impact sont suffisantes et que la priorité doit porter sur l'évaluation des textes adoptés La qualité d'une étude d'impact ne préjuge pas la qualité de la loi : il peut y avoir de mauvaises études d'impact et de bonnes lois ; il peut aussi y avoir de très belles études d'impact et des lois insatisfaisantes. Il faut admettre qu'il s'agit là d'un exercice difficile : comment juger les effets d'une disposition encore inexistante ? J'ajoute, à l'attention de M. le sénateur Montaugé et du groupe socialiste et républicain, en anticipant un peu sur nos débats de l'après-midi, que le défi serait encore plus difficile à relever avec une étude d'impact plus « qualitative ». Il est déjà délicat de satisfaire les parlementaires avec des critères dits « quantitatifs ceux actuellement requis : qu'en serait-il avec des critères plus souples et qui se définissent encore moins facilement ? Il faut, à cet égard, se rappeler que le Conseil constitutionnel se garde, avec raison, de définir ce que serait une étude d'impact satisfaisante. Saisi par le Premier ministre à l'occasion de l'examen du projet de loi NOTRe, le Sénat refusant d'inscrire le texte à l'ordre du jour au motif que son étude d'impact ne respectait pas les prescriptions de la loi organique, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que les dispositions organiques n'avaient pas été méconnues, alors que les critiques étaient féroces. En réalité, lorsque nous élaborons la loi, nous ne manquons pas d'analyses ou d'études, ni même de l'avis d'organismes indépendants, qui ne se privent nullement de le donner. Nous manquons souvent de suite dans les idées. Nous devrions pouvoir prendre le temps de mieux évaluer la loi et d'en tirer les leçons quant à sa pertinence, à son efficacité ou à son utilité. Plutôt que de nous livrer, toujours plus avant, à un exercice d'analyse qui, quelles que soient les garanties qui l'entourent, sera toujours frustrant, nous devons consacrer des moyens importants à l'évaluation et au contrôle des politiques publiques. Nous devons, pour cela, donner au Parlement un « droit de suite » : le droit de légiférer sur la base de ses propres évaluations.

Le Président de la République et le Premier ministre ont plusieurs fois évoqué un « printemps de l'évaluation », par exemple avec un examen rénové de la loi de règlement, mais aussi- cette piste a été envisagée devant la Cour des comptes -avec l'audition de chacun des ministres par les commissions parlementaires sur le bilan de l'année écoulée et sur le programme de travail de l'année à venir. Il faudrait, en somme, que le Gouvernement passe moins de temps à convaincre, et plus à rendre compte. Cela vaut en matière budgétaire, bien sûr, comme pour les autres domaines de l'action publique. Le Gouvernement doit se rendre disponible pour présenter au Parlement les résultats ministériels, tant dans l'application des lois que dans la performance des politiques publiques. C'est une ambition forte, et le gage d'un fonctionnement sain de notre démocratie et de la séparation des pouvoirs. Rééquilibrer le calendrier parlementaire, en somme, tel est l'enjeu pour nous. Cela passera peut-être, aussi, par l'enrichissement de la semaine de contrôle, qui n'apporte aujourd'hui pas pleinement satisfaction aujourd'hui aux parlementaires, alors qu'elle pourrait être un outil formidable de suivi et de contrôle de l'action du Gouvernement. De tout cela, mesdames, messieurs les sénateurs, vous serez amenés à discuter à brève échéance. C'est une position de principe ambitieuse, une volonté forte du Gouvernement et du Président de la République, qui seront soumises à votre examen dans les semaines et les mois à venir. Des consultations vont être engagées à partir de cette semaine pour recueillir les avis et les expertises de toutes les parties prenantes en vue de la révision constitutionnelle, qui devra être adoptée avant l'été. Cette proposition de loi organique vient donc heurter le calendrier de cette grande réforme constitutionnelle. Cela justifie les plus grandes réserves du Gouvernement quant à son éventuelle adoption. En second lieu, le Gouvernement émet sur ce texte plusieurs réserves d'ordre juridique qui plaident également pour un rejet. Sans trop anticiper le débat sur chacun des amendements, je soulignerai d'ores et déjà que ces réserves portent principalement sur l'article 2 de la proposition loi, qui prévoit que les évaluations figurant dans les études d'impact « sont également réalisées par des organismes indépendants ». Cette rédaction convient mieux au Gouvernement que la version initiale du texte, qui prévoyait le recours à des organismes publics indépendants et pluralistes, ainsi qu'à des personnalités qualifiées désignées par le Parlement, pour la réalisation des évaluations figurant dans les études d'impact. Elle lève ainsi la principale objection qui pouvait être formulée à l'égard du texte initial, tenant au fait qu'une étude d'impact a pour objet de compléter l'exposé des motifs des projets de loi par une analyse précise des avantages attendus et des multiples incidences du texte. Une étude d'impact ne constitue donc pas un diagnostic préalable pouvant relever de la seule compétence d'une autorité indépendante. Néanmoins, l'obligation de contre-expertise indépendante que ces dispositions entraînent pourrait ne pas être conforme aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Cet article n'habilite en effet le législateur organique qu'à réglementer les conditions de « présentation » des projets de loi. Or une telle exigence pourrait être regardée comme touchant non pas à la présentation, mais à l'élaboration même des projets de loi. projets de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà des réserves d'ordre juridique que j'ai brièvement mentionnées et sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir lors de l'examen des amendements, vous aurez compris que ce sont des raisons de principe, de calendrier et d'orientations de la révision constitutionnelle qui conduiront le Gouvernement à donner un avis défavorable à l'adoption de la présente proposition de loi organique par votre assemblée. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur de la commission des lois, monsieur l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, dans le rapport pour « une VRépublique plus démocratique », le comité de réflexion présidé par Édouard Balladur recommandait « que l'existence de ces études d'impact soit une condition de la recevabilité d'un projet de loi à charge pour le Conseil constitutionnel de vérifier [ ...] que ce document satisfait aux exigences qu'une loi organique pourrait prévoir ». Cette conception, très clairement énoncée, a guidé le pouvoir constituant en 2008 lors de la modification de l'article 39 de la Constitution, puis lors de l'adoption de la loi organique du 15 avril 2009. Cela n'a pas Cela n'a pas empêché la pratique et la jurisprudence constitutionnelle de s'éloigner de l'esprit du texte de 2009. Dès les premières manifestations de cette dérive, le groupe du RDSE avait réagi en proposant de clarifier la rédaction de l'article 8 afin que les dispositions de celle-ci ne puissent plus donner lieu à une interprétation trop restrictive, aboutissant au contrôle, minimal, de la simple existence d'une étude d'impact. Si le législateur avait fixé des critères, c'était pour que le Conseil constitutionnel en sanctionne le cas Le caractère imparfait des études d'impact est aujourd'hui largement reconnu, y compris par le Conseil d'État. Nous saluons donc l'initiative prise par nos collègues socialistes de remettre ce sujet à l'ordre du jour, ainsi que les améliorations apportées par le rapporteur, dans le prolongement des réflexions conduites par notre collègue François Pillet. La généralisation des études d'impact à tous les projets de loi n'a pas produit les effets escomptés, à savoir l'amélioration de la qualité de la loi et la limitation de l'inflation normative, leur qualité étant trop aléatoire. Certains d'entre nous gardent le souvenir de l'étude fournie à l'appui de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et qui n'expliquait ni les calculs retenus, ni le détail des options possibles, ni les raisons pour lesquelles certains découpages avaient été préférés à d'autres. Dans de nombreux cas, les études d'impact donnent l'impression d'être destinées à noyer leurs lecteurs sous des détails encyclopédiques, sans pour autant répondre à l'objectif fixé par la loi organique. Soumettre aux parlementaires des études d'impact de qualité est également un enjeu en termes de rééquilibrage institutionnel, dans un contexte de marginalisation du Parlement. L'avenir du parlementarisme en France dépend de la possibilité, pour les membres de nos assemblées, de disposer de données agrégées pour formuler des propositions réalistes,

Bien que les modifications proposées ne permettent pas de renforcer le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur le contenu des études d'impact, je me félicite du consensus trouvé sur ce texte en commission. Cela a permis d'étoffer la proposition de loi. Si quelques membres du groupe regrettent que la réflexion de notre collègue Montaugé sur les nouveaux indicateurs de richesse ne soit pas prise en compte dans la version finale, nous sommes en revanche très favorables à l'extension de la liste des informations devant figurer dans l'étude d'impact. Il s'agit, en particulier, d'y inclure les données concernant les collectivités territoriales et les entreprises, au travers de l'article 1 A, et les données relatives aux moyens humains et informatiques nécessaires à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions, au travers Est également reprise l'obligation de préciser « l'apport des dispositions envisagées en matière de simplification et, en cas de création d'une nouvelle norme, les normes dont l'abrogation est proposée ». Cela permettra d'atteindre l'objectif de simplification des normes cher à l'ensemble des membres du groupe RDSE.

Si nous nous réjouissons de cet apport, nous serons néanmoins attentifs aux modalités de désignation de ces organismes, ainsi qu'aux les modalités de réalisation de ces évaluations, dans un souci de transparence, le texte ouvrant la voie à l'évaluation par des organismes privés. L'alinéa 2 permettant, le cas échéant, la prise en compte des avis rendus par le Conseil national de l'évaluation des normes représente une réelle avancée, car cela permettra d'estimer par avance les coûts d'une mesure, non seulement pour nos collectivités territoriales, mais également pour nos entreprises. disposition aurait pu s'avérer bien utile pour nombre de dirigeants d'exécutifs locaux lors des différentes réformes de ces dernières années. L'allongement des délais de saisine du Conseil constitutionnel par la conférence des présidents pourrait également aller dans le bon sens si elle s'accompagnait d'une évolution effective du contrôle assuré par le Conseil

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je voudrais moi aussi saluer cette proposition de loi visant à améliorer la qualité des études d'impact

en déplorant « l'absence de contrôle externe sur la qualité de l'étude d'impact, faite par l'administration qui prépare la norme », « l'absence de confrontation systématique

seul projet de décret relatif aux obligations de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

plus large, quel travail législatif voulons-nous pour demain ? Quelle confiance notre pays place-t-il en ses parlementaires ? Le sujet dont nous débattons cet après-midi fait naturellement écho- cela a été dit -à la réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la République. Or, en la matière, les signaux envoyés par l'exécutif sont extrêmement préoccupants. Je pense à deux mesures visant à restreindre le droit d'amendement qui font la une des journaux d'aujourd'hui : l'interdiction du dépôt en séance publique d'un amendement ayant été rejeté par la commission chargée d'examiner le texte en amont ; la limitation, au prorata de la taille du groupe, du nombre d'amendements pouvant être déposés par un parti d'opposition. Ces mesures reviennent sur un droit constitutif du Parlement : ce n'est pas acceptable. Je ne partage pas cette vision du travail parlementaire et du rôle du Parlement. Au contraire, je crois au courage politique et au caractère

que le temps parlementaire est trop long, que mener des auditions et associer le plus en amont possible les parties prenantes, faire se confronter les points de vue, débattre entre représentants de sensibilités politiques différentes dans cet hémicycle, y compris à une heure avancée de la nuit,

Oserais-je dire que le temps consacré par un parlementaire moyen à la lecture de l'étude d'impact, qui représente souvent des centaines de pages, avant qu'il ne se prononce

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quand on se rappelle avec quelle désinvolture le Conseil constitutionnel a validé l'étude d'impact accompagnant le projet de redécoupage régional, on a quelques doutes sur la destinée des propositions d'amélioration desdites études que pourraient faire les parlementaires ... D'ailleurs, le Gouvernement vient de nous le dire, tout va très bien

Nous y reviendrons. C'est fou comme, ces derniers temps, les propositions de loi ont tendance à rétrécir au lavage de la commission des lois ! Là encore, je m'interroge sur l'effet réel de la réforme constitutionnelle de 2008.

2015, ou loi Sas. Comme on sait, il s'agit notamment d'indicateurs d'inégalités, de qualité de vie, de développement durable et, d'une manière générale, d'indicateurs qualitatifs. Ils auraient été très utiles lors de l'examen de la loi NOTRe ! Notre « mission

que « le renforcement de certaines collectivités au détriment d'autres a généré des gagnantes et des perdantes qui ont le sentiment d'être des oubliées de l'État, notamment les petites communes rurales Avec la multiplication des métropoles, on risque d'en avoir une cruelle confirmation. Quand on sait, en outre, comment est fabriqué le PIB, qui laisse délibérément de côté la plupart des activités non marchandes, mais qui intégrera bientôt le trafic de drogue, on a tout lieu de soutenir cette proposition ! La seconde disposition intéressante à mes yeux tendait à ce que ces études d'impact ne soient plus « mitonnées

des points et des sujets qu'elles souhaitent voir traiter dans l'étude d'impact. Je ne suis pas le seul à avoir constaté que les études d'impact répondent rarement aux interrogations des parlementaires : on y trouve

par les amendements qu'il a déposés avec son groupe, nous soutiendrons le rétablissement de l'article 1er, supprimé par la commission- on se demande bien pourquoi ! -, ainsi que le rétablissement du caractère public des organismes indépendants chargés de réaliser l'étude d'impact. Nous ne pensons pas, en effet, qu'être soumis aux contraintes du marché et au bon vouloir de ses clients soit la meilleure garantie d'indépendance ... Nous avons proposé, en outre, que les amendements déposés par le Gouvernement

dans lequel nous abordons la discussion des deux textes soumis à notre examen, en regrettant que la commission ait cru bon de transformer une proposition de loi simple, claire et utile en un texte trop compliqué pour avoir une chance de survivre à la navette. Mais peut-être était-ce le but

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui nous invite à dresser un bilan du recours aux études d'impact.

en intégrant dans les études d'impact l'évaluation des conséquences, pour les entreprises et les collectivités territoriales, notamment en termes de coût, des dispositions envisagées. Il y ajoute l'évaluation des moyens humains, financiers et informatiques nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi qu'une analyse du bilan des normes créées et abrogées. Par ailleurs, il propose le recours à un certain nombre d'organismes indépendants énumérés de manière non limitative, en complément du débat,

sur la révision constitutionnelle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la conférence des présidents de l'assemblée pourrait constater que les obligations relatives aux études d'impact ne sont pas remplies.

du groupe de travail sénatorial sur la révision constitutionnelle. Je le dis immédiatement, ces propositions ont l'agrément du groupe Union Centriste. Cela étant,

s'agissant des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, des évaluations préalables qui en tiennent lieu -a constitué une réelle amélioration, puisqu'en principe elle oblige, depuis 2009, le Gouvernement à éclairer à éclairer le Parlement sur les raisons de légiférer, sur les options alternatives et sur l'ensemble des conséquences des dispositions envisagées. La proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui prévoit, d'une part, que les études d'impact des projets de loi doivent comporter une « évaluation qualitative de l'impact des dispositions envisagées au regard des nouveaux indicateurs de richesse et, d'autre part, que les évaluations devant figurer dans les études d'impact doivent être réalisées par des « organismes publics indépendants et pluralistes », auxquels les assemblées parlementaires pourraient adjoindre des personnalités qualifiées. L'examen de ce texte renvoie au débat sur l'utilité et sur la qualité des études d'impact, alors que le Gouvernement, conformément à l'annonce faite le 3 juillet 2017 par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, élabore un projet de révision constitutionnelle dont la discussion pourra précisément être l'occasion d'évoquer d'évoquer la question de la qualité des études d'impact. L'obligation de joindre aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d'État, puis lors de leur dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre des deux assemblées, une étude d'impact comportant une série d'informations et d'évaluations, a été instaurée par la loi organique du 15 avril 2009. Cette obligation d'information du Parlement à la charge du Gouvernement est entrée en vigueur pour les projets de loi déposés à compter du 1 septembre 2009.

En effet, la pratique s'est révélée décevante depuis 2009 au regard des espoirs placés dans cet outil pour faire progresser la qualité du processus d'élaboration des lois. C'est pourquoi l'examen de cette proposition de loi organique est l'occasion de reprendre les travaux antérieurs du Sénat sur les études d'impact et d'introduire dans le texte les propositions formulées en janvier 2018 par le groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, lorsqu'elles ne nécessitaient pas de modification de la Constitution. Je me réjouis donc que la commission des lois, sur l'initiative du rapporteur, ait décidé- à l'unanimité -de relever le niveau d'exigence pour les études d'impact des projets de loi, par le biais de l'adoption de sept amendements. Ainsi, en complément des évaluations réalisées par le Gouvernement, les études d'impact devront comporter des évaluations réalisées par des organismes indépendants, afin de renforcer l'objectivité de l'information du Parlement sur les conséquences des projets de loi. Les études d'impact devront aussi comporter une évaluation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des projets de loi par l'État et les administrations publiques, d'un point de vue à la fois humain, budgétaire et informatique, ainsi que des délais nécessaires à leur mise en oeuvre. En outre, elles devront évaluer spécifiquement les coûts induits par les projets de loi pour les collectivités territoriales et pour les entreprises, ainsi que l'apport des projets de loi en matière de simplification. Elles devront également préciser, dans l'hypothèse où la création de nouvelles normes est envisagée, les normes qu'il est proposé d'abroger en contrepartie. Les avis rendus par le CNEN devront ainsi y être joints. Enfin, en matière de procédure, la conférence des présidents de la première assemblée saisie devra disposer d'un délai allongé de dix à trente jours pour apprécier la qualité de l'étude d'impact et s'opposer à l'inscription à l'inscription du projet de loi concerné à son ordre du jour si l'étude d'impact est jugée insuffisante. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les amendements adoptés en commission des lois modifient de façon substantielle la proposition de loi organique en y incorporant les conclusions du groupe de travail sur la révision constitutionnelle.

de nos décisions, sans pour autant que nous abdiquions nos convictions de gauche, de droite ou d'ailleurs

fins d'amélioration de la qualité de la loi et de limitation de l'inflation législative, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 15 avril 2009 ont instauré l'obligation de joindre aux projets de loi une étude d'impact comportant une série d'informations et d'évaluations. L'étude d'impact a un rôle : éclairer le Parlement. Toutefois, comme l'a souligné notre rapporteur, qu'il faut remercier de son travail, les études d'impact ont fait l'objet de critiques régulières et parfois sévères quant à leur utilité, à leur contenu et à leurs modalités d'élaboration. Tantôt pures formalités, tantôt justifications d'un projet de loi, elles ne donnent pas satisfaction et ne permettent pas de fournir une information de qualité au Parlement.

La proposition de loi organique porte, d'une part, sur le contenu des études d'impact, et, d'autre part, sur la nature des organismes qui peuvent les réaliser.

sur le PIB, parce que cette grille d'interprétation conditionne notre façon d'appréhender le monde, et donc la manière dont sont conduites les politiques publiques. Si le PIB est un indicateur indispensable pour mesurer la croissance, voire pour juger de l'efficacité des politiques publiques, il n'est pas, il ne peut plus

des Nations unies, avec l'IDH, l'indicateur de développement humain, ou de l'OCDE, de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi ou encore de France Stratégie.

Il est donc nécessaire pour nous d'embrasser l'ensemble des disciplines, de développer des indicateurs alternatifs, afin de mesurer vraiment la qualité de la décision publique.

les dix indicateurs dont nous disposons sont « un outil unique. C'est un constat sans appel de l'évolution de notre société, c'est un rappel puissant au Parlement et au Gouvernement de leurs responsabilités.

la réalisation d'évaluations complémentaires par des organismes indépendants, dont le contenu serait intégré au document rendant compte de l'étude d'impact. Nous pouvons nous féliciter de cette avancée, qui permettra de renforcer l'objectivité de

pour apprécier la qualité de l'étude d'impact et s'opposer, s'il y a lieu, à l'inscription de l'examen du projet de loi à son ordre du jour. Nous approuvons l'ensemble de ces propositions, qui concourront à améliorer la qualité et l'objectivité des études d'impact et à enrichir notre culture de l'évaluation. Nous voterons bien entendu l'évaluation. Nous voterons bien entendu cette proposition de loi organique, mais nous estimons, comme notre collègue Franck Montaugé, que la réflexion sur les nouveaux indicateurs de richesse doit être poursuivie et que ces indicateurs mériteraient d'être intégrés dans nos grilles d'interprétation

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la révision constitutionnelle de 2008 a introduit une nouvelle procédure législative à l'article 39 de la Constitution.

Les études d'impact doivent servir à la fois deux objectifs : relever les effets de la législation en vigueur que l'on envisage de modifier, et anticiper les effets des modifications apportées par le projet de loi à cette législation. Pour être valables, elles doivent satisfaire à neuf obligations définies par la loi organique. Elles ont pour objets essentiels de répondre au problème de l'inflation législative, en faisant état des lois existantes, et d'anticiper les difficultés auxquelles sera confronté le législateur, notamment l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus de la mise en oeuvre des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques ou morales intéressées.

Si cette proposition de loi répond à des objectifs louables, sa discussion intervient alors même que l'application de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 reste tout à fait partielle et insatisfaisante pour le Parlement.

Cette situation a été clairement mise en évidence lors de l'examen du projet de loi NOTRe, en 2014. À l'unisson, plusieurs groupes politiques du Sénat avaient déploré les lacunes de l'étude d'impact accompagnant ce projet de loi. La conférence des présidents avait entériné ce constat et décidé de retirer le texte de l'ordre du jour. Malgré cette décision, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, avait jugé que le texte avait été présenté dans des conditions conformes à la loi organique, et s'était déclaré impuissant à juger la qualité de l'étude d'impact. Il est évident qu'une modification de la loi organique s'impose, afin de rendre indispensable la réalisation d'une étude d'impact reposant sur des indicateurs précis, dont la qualité pourra être appréciée par le Conseil constitutionnel.

%. En juillet dernier, le Premier ministre annonçait vouloir supprimer deux normes pour toute nouvelle norme créée ; il est temps de se saisir de ces questions, depuis longtemps évoquées mais jamais traitées. Cette proposition de loi nous permet également d'échanger sur l'application de l'article 39 de la Constitution et de pointer du doigt les défaillances de la législation actuelle concernant la réalisation et l'examen de ces études d'impact. Il est de notre intérêt de revoir en profondeur la manière dont celles-ci sont réalisées et examinées. Elles doivent, à mon sens, permettre au Parlement de statuer sur une loi sur le fondement d'une connaissance approfondie des dispositions de celle-ci. Les neuf obligations inscrites dans la loi organique n'ont pas de valeur si elles ne sont pas correctement respectées et si le Conseil constitutionnel n'a aucun pouvoir pour contester la qualité

d'un Parlement fort. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

C'est pourquoi je m'interroge sur l'opportunité d'en étendre le champ et d'en élargir le contenu, comme le propose notre collègue. Est-il nécessaire de préciser, mes chers collègues, au bout du compte, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des entreprises, ce sont bien les Français qui supportent les coûts de l'inflation normative ? Dans ces conditions, quel bénéfice y aurait-il à prendre en compte des indicateurs de richesse si cela ne permet pas d'améliorer le contenu des projets de loi ?

et que cela a un impact très significatif sur l'emploi. En tant que membre de la délégation sénatoriale aux entreprises, je veux d'ailleurs faire référence à l'excellent rapport d'information de nos collègues Élisabeth Lamure et Olivier Cadic intitulé « Simplifier efficacement pour libérer les entreprises ».

C'est pourquoi, si nous devons revoir ce dispositif, je souhaite, pour ma part, que cette révision le rende plus efficient, afin que ces études d'impact soient utiles au travail législatif, mais aussi moins pénalisantes pour le secteur économique. améliorer la qualité des études d'impact est certes louable, il faut aussi introduire, si nous voulons tendre réellement vers l'objectif ambitieux d'une simplification réglementaire et administrative,

Dans un monde qui évolue très rapidement, dans une économie mondialisée, il faut évaluer en toute objectivité les politiques mises en oeuvre, sans esprit partisan, à l'aide d'éléments factuels. pas craindre une évaluation approfondie des résultats obtenus au regard des objectifs fixés aux lois, bien au contraire. Pour renforcer le rôle du Parlement, il est utile d'évaluer les lois qui ont été votées. Je suis donc réservée sur la pertinence de ce texte, qui ne nous permettra pas d'améliorer les règles. À l'heure où les Français demandent une véritable simplification et davantage de lisibilité, il est grand temps d'améliorer l'efficience des études d'impact.

Franck Montaugé. Il est dommage que, en supprimant l'article 1 de ce texte, la commission n'ait pas voulu prendre en compte la question importante de la pertinence des indicateurs utilisés dans les études d'impact. dans les études d'impact. Cela a été rappelé, la commission Stiglitz a relancé le débat sur les indicateurs de richesse et sur l'intégration d'objectifs de développement durable dans les politiques publiques,

la question, pour nous parlementaires, est de savoir comment articuler, de façon cohérente et lisible, les objectifs de développement durable auxquels notre pays a souscrit et les indicateurs dont nous disposons pour la réalisation des études d'impact et, plus largement, l'évaluation des politiques publiques.

il s'agit d'un problème très concret. J'ai évoqué tout à l'heure la loi NOTRe, je pourrais évoquer toutes les lois de réforme territoriale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

Selon le critère du poids de la réglementation, la France est classée au 115 rang sur 138 pays par le Forum économique mondial. De nombreux pays européens ont bien compris l'enjeu en termes de compétitivité plusieurs d'entre eux avant d'adopter le rapport d'information intitulé « Simplifier efficacement pour libérer les entreprises ». Les préconisations de ce rapport nous ont conduits à déposer, en septembre dernier, plusieurs textes cosignés par de nombreux membres de la délégation, dont deux propositions de loi : une proposition de loi organique prévoyant que l'étude d'impact mentionne les conséquences du projet de loi en termes de simplification du droit, afin d'inciter le Gouvernement à mieux prendre en compte cet impératif- je me réjouis que la commission des lois ait intégré cette disposition dans son texte -et une proposition de loi constitutionnelle visant à introduire une obligation de compenser la création de toute nouvelle charge pour les entreprises par la suppression d'une charge équivalente. Dans le même esprit, l'article 1 du présent texte pose le principe de l'abrogation de normes

en garantissant que la charge financière que représente la norme abrogée l'emporte sur celle de la norme créée. Nos voisins Allemands, en procédant ainsi, sont parvenus à économiser 14 milliards d'euros en cinq ans. La France doit pouvoir réussir elle aussi à alléger enfin le boulet qui freine ses entreprises dans la course mondiale

en matière de simplification et, en cas de création d'une nouvelle norme, les normes dont l'abrogation est proposée. Pour garantir que cette avancée sera substantielle, il convient d'assurer que la simplification normative apporte un allégement effectif, ce qui implique que la charge financière engendrée par les normes nouvellement créées soit inférieure à la charge financière représentée par les normes supprimées En janvier 2016, le Sénat a adopté une proposition de loi constitutionnelle qui prévoyait déjà d'assortir toute mesure législative ou réglementaire ayant pour effet de créer ou d'aggraver une charge pour les collectivités territoriales de la suppression de mesures représentant une charge équivalente

Elle est peut-être redondante avec ce que la loi organique prévoit déjà, à savoir la mention des coûts et bénéfices attendus. C'est pourquoi la commission

l'article ne revêtirait qu'une portée résiduelle, dans la mesure où l'impact sur l'ordre juridique interne mais également l'incidence économique d'une mesure législative doivent déjà être précisés dans les études d'impact, sur le fondement de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. À l'inverse, si le dispositif de l'amendement devait être interprété de manière beaucoup plus contraignante,

sur l'article. L'article 2 de la proposition de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les études d'impact telles que prévues par la loi organique de 2009 soient réalisées par des organismes publics indépendants et pluralistes. La commission des lois a jugé nécessaire d'étendre aux organismes privés la possibilité de réaliser ces évaluations. Or nous considérons, pour notre part, que c'est le caractère public de ces organismes qui garantit leur indépendance, en empêchant d'éventuels conflits d'intérêts liés notamment au mode de financement des organismes privés. L'amendement vise donc à réintroduire le texte initial de la proposition de loi, qui prévoyait que les évaluations des conséquences économiques, sociales, financières et environnementales des projets de loi puissent être réalisées par des organismes publics indépendants.

En effet, à la fin des années soixante-dix, des rapports publics avaient dénoncé de manière récurrente le monopole que détenait l'administration dans le domaine de l'expertise économique et sociale. Le rapport de René Lenoir et de Baudouin Prot, commandé par Valéry Giscard d'Estaing en 1979, a joué un rôle extrêmement important dans la démocratisation de l'analyse économique et sociale en France.

publiques, assurent « le pluralisme dans l'analyse économique, l'évaluation des politiques publiques et l'étude de la conjoncture économique, en France et en Europe », comme l'indiquent les statuts de l'OFCE.

Je propose donc, mes chers collègues, que les différentes versions des projets de loi et les éventuelles saisines rectificatives soient jointes à l'étude d'impact. Lors de l'examen de l'avant-projet, le Conseil d'État dispose de l'étude d'impact et ne manque pas de s'appuyer sur elle pour rendre son avis.

Il est également proposé que l'avis du Conseil d'État soit lui aussi annexé à l'étude d'impact et ainsi rendu public. Dans les faits, ses avis sont rendus publics depuis la fin du précédent quinquennat. Il est donc proposé d'officialiser cette pratique en l'inscrivant dans la loi, tout en permettant au Gouvernement de s'opposer à cette publication intégrale pour des motifs impérieux d'intérêt général. L'avis serait alors remplacé par une note synthétisant les principales observations. Si l'avis du Conseil d'État devait être publié officiellement, il serait fort logique que l'avant-projet l'accompagne. Plus généralement, mes chers collègues, j'avais souhaité profiter de cette initiative parlementaire pour modifier d'autres dispositions relatives à nos travaux, mais l'irrecevabilité de mes amendements m'a été opposée en commission. En quelques mots, sans remettre en cause leur droit d'amendement, je considère que le Gouvernement et la commission saisie au fond devraient être soumis aux mêmes délais de dépôt que les parlementaires, sauf pour leurs amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. De même, le Gouvernement pourrait être tenu de réaliser une étude d'impact pour ses amendements. En effet, il a aujourd'hui trop souvent tendance à s'exonérer de à s'exonérer de ses obligations en insérant des dispositions nouvelles par voie d'amendement, donc sans avis du Conseil d'État ni réalisation d'une étude d'impact. De surcroît, ces amendements ne sont souvent déposés que quelques minutes avant la séance ... Il s'agit là, mes chers collègues, de propositions dont nous débattrons lors de la révision constitutionnelle,

traditionnellement, ceux-ci ne sont pas rendus publics et ne sont pas communicables aux personnes qui en font la demande, car ils entrent dans la catégorie des documents administratifs dont la consultation et la communication porteraient atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, tel que défini par le 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application d'une décision orale du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015 lors de la cérémonie des voeux aux corps constitués, les avis sur les projets de loi sont, depuis le 19 mars 2015, intégralement rendus publics par le Gouvernement sur le site Légifrance dès que ces textes ont été délibérés en conseil des ministres. Le Gouvernement les transmet à la première assemblée saisie au moment du dépôt du projet de loi. Le texte retenu par le Conseil d'État, quant à lui, n'est pas rendu public. Par exception, cette nouvelle pratique ne s'applique pas aux avis sur les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale ou de ratification d'une ordonnance ni aux avis sur les projets de loi autorisant la ratification d'un engagement international. Nous considérons que cette pratique, décidée par l'exécutif en 2015, permet d'assurer un juste équilibre entre la préservation du rôle du Conseil d'État en tant que conseil du Gouvernement

Comment voulez-vous, dans ces conditions, aboutir à un accord en commission mixte paritaire ? C'est pourquoi l'absence de règles limitant la possibilité, pour la seconde assemblée saisie,

groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être, présentée par M. Franck Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain Dans la discussion générale, la parole est à M. Franck Montaugé, auteur de la proposition de loi organique.

améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi, le texte dont nous allons maintenant discuter a aussi pour objet d'améliorer la fabrique de la loi à partir de l'implication effective et structurée des parlementaires dans le processus d'évaluation des politiques publiques. L'article 24 de la Constitution donne explicitement au Parlement la mission d'évaluer les politiques publiques. Les missions d'enquête, les rapports d'information y concourent, les études d'impact abordent le sujet, mais aucune démarche ou organisation, propre à chaque chambre ou commune, n'est prévue dans la loi ou dans les règlements intérieurs des assemblées. Les politiques publiques et leur évaluation constituent un champ de savoir et de recherche à part entière. Cette « science de l'État en action », comme certains l'appellent, est aussi la branche la plus récente de la science politique. Si tous les acteurs de la société sont concernés de manière générale, au titre de leur citoyenneté, ils le sont aussi en tant qu'acteurs et sujets de politiques publiques sectorielles, spécifiques

Au-delà de l'appréciation personnelle que chacun d'entre nous porte sur son expérience parlementaire, la question de l'efficacité, si ce n'est de l'efficience, de notre action collective et de notre contribution aux évolutions de la société française est posée dans le débat public.

C'est là tout le sens et la raison d'être de ce texte. Les expériences antérieures de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, l'OPEL, de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, l'OPEPP, et même de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois n'ont pas été probantes. Forts de ce constat, nous avons voulu, au travers de ce texte, complémentaire du précédent, faire des propositions visant à nous doter d'une démarche structurée à même de permettre aux parlementaires de monter en connaissance et en compétence sur le sujet, à la fois politique et technique, de l'évaluation des politiques publiques. Ma conviction est que, en travaillant en lien avec les institutions spécialisées et le monde académique compétent sur ces sujets, en nous appuyant également sur les compétences et l'expertise remarquable des administrations

les politiques publiques sont le lieu où des sociétés définissent leur rapport au monde et à elles-mêmes ; une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action gouvernementale dans un secteur de la société ou un espace géographique. Quant à l'évaluation, c'est l'activité de rassemblement, d'analyse et d'interprétation de l'information concernant la mise en oeuvre et l'impact de mesures visant à agir sur une situation sociale, ainsi que la préparation de mesures nouvelles.

assistée d'un conseil scientifique pluraliste, composé de trente membres- économistes, sociologues, historiens, anthropologues ... -désignés pour trois ans, dans le cadre du règlement de la délégation. ce conseil serait d'informer le Parlement sur les conséquences des politiques publiques sur le bien-être et sur leur soutenabilité, de mettre en oeuvre et d'animer une plateforme participative numérique relative aux nouveaux indicateurs de richesse-

L'article 3 prévoit qu'une contre-expertise indépendante du rapport prévu par la loi Sas soit réalisée en vue de favoriser l'objectivité de l'évaluation des politiques publiques portée au débat public, les organismes chargés de conduire cette étude étant désignés tous les deux ans par décret en Conseil d'État. Des membres éminents de la commission des lois estimant que le dispositif présenté est trop lourd, trop complexe, le rapporteur proposera dans quelques instants le renvoi du texte à la commission, pour préserver la suite de la réflexion.

que la chambre haute s'engage sur la voie de l'évaluation des politiques publiques dans le cadre d'une adaptation de son règlement intérieur donnant aux commissions toutes prérogatives en la matière. Toutefois, je tiens à attirer l'attention sur un point qui me paraît fondamental

Il nous faudra bien envisager, à certains moments et sur certains sujets, d'entreprendre un travail commun, à l'aune des grands enjeux devant constituer le substrat, le postulat de nos raisonnements et de nos méthodes d'évaluation.

La complexité de nos sociétés affecte nos politiques publiques. Il nous faudra donc trouver une organisation interne adaptée pour tenter d'appréhender cette complexité du réel

C'est aussi pour cette raison que les nouveaux indicateurs de richesse tiennent une place importante dans notre texte et que nous souhaitons que leur pertinence soit évaluée et qu'ils puissent faire l'objet d'évolutions dûment documentées.

telles que le FMI et l'OCDE et des institutions moins orthodoxes -, nous pensons que la question des inégalités doit faire l'objet d'un suivi particulier, régulier, et que le Sénat, qui se veut défenseur des libertés, doit donner l'exemple en la matière.

pour terminer, aborder la dimension démocratique de l'évaluation des politiques publiques. L'analyse des politiques publiques doit nous permettre, au-delà des valeurs et des options partisanes qui sont les nôtres, de porter un autre regard sur le politique. Le modèle d'action Le modèle d'action publique de la France a connu, depuis le XIX siècle, des transformations profondes. Le mode d'action publique issu de l'après-guerre, qui s'est développé jusque dans les années soixante-dix, était construit sur le rôle central de l'État en matière de développement économique. L'élite politico-administrative de cette période avait développé les politiques publiques à partir d'un modèle fondé sur la place centrale de l'État dans le développement économique. La place grandissante de l'Union européenne et l'ouverture à une économie de plus en plus mondialisée ont, petit à petit, débouché sur un affaiblissement de la centralité de l'État. La disqualification, voire le rejet, du politique-

chercheur honoraire au CNRS et spécialiste des politiques publiques, « cette crise [ ...] débouche sur une profonde transformation de l'espace public, entendu à la fois comme lieu de production du sens et comme lieu d'expression des intérêts sociaux en même temps qu'à l'émergence de nouveaux rapports sociaux entre l'individu et l'action collective ». ». Il ajoute que cette crise « doit surtout conduire à réfléchir sur la fonction politique aujourd'hui et notamment au découplage croissant entre la fonction d'élaboration des politiques publiques () et la fonction de représentation politique politique (). [ ...] Entre les contraintes liées au contexte extérieur qui déterminent de plus en plus clairement le contenu des politiques publiques et les demandes de nouvelles formes de participation politique formulées par les citoyens, les responsables politiques devront trouver de nouveaux modes de transaction sous peine de voir se développer les différentes formes de populisme porteuses de visions du monde à la fois simplistes et dangereuses. » La révision constitutionnelle aurait pu être posée en ces termes.

mais aussi de suivre scrupuleusement ses conditions d'application ou de non-application, à commencer par la publication des textes réglementaires.

l'examen de cette proposition de loi nous permet de prolonger le débat entamé au travers de nos échanges sur la proposition de loi organique, et en particulier sur la pertinence du recours aux nouveaux indicateurs de richesse prévus dans la loi Sas. Si le sort de cette proposition de loi, sans préjuger le vote de votre assemblée, semble ne pas faire de doute- la commission ayant une nouvelle fois déposé une motion tendant à son renvoi à la commission -, son examen représente, pour le Gouvernement et le Parlement, l'occasion de réfléchir ensemble aux formes que pourrait prendre la mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. La présente proposition de loi vise en effet « à favoriser le développement de nouveaux indicateurs de richesse, leur utilisation et leur appropriation citoyenne afin de faire rentrer dans les moeurs une autre culture de l'évaluation fondée sur des indicateurs alternatifs au PIB À ce titre, elle tend à enrichir la loi du 13 avril 2015, qui se borne à prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur ce sujet. Ce texte prévoit la création d'une délégation parlementaire dénommée « conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être », sur le modèle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et technologiques, chargée « d'informer le Parlement sur la politique suivie par le Gouvernement, notamment en matière de choix budgétaires, au regard de nouveaux indicateurs de richesse ». La proposition de loi prévoit également que ce conseil parlementaire évalue, tous les trois ans, la pertinence desdits indicateurs de richesse prévus par la loi Sas et formule des propositions. Enfin, le texte précise que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de la loi Sas doit faire l'objet d'une contre-expertise par un ou plusieurs organismes indépendants. Ce texte soulève en somme deux questions : comment doit s'organiser l'évaluation des politiques publiques ? Sur quels critères doit-elle s'appuyer pour être pertinente ? La première La première question rejoint les réflexions dont je vous ai fait part tout à l'heure lors de mon intervention liminaire sur la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi. La volonté du Gouvernement et du Président de la République est de donner au Parlement tous les outils pour renforcer ses méthodes d'évaluation des lois, ses capacités d'expertise des effets emportés par les dispositions votées et pour remplir au mieux sa mission de contrôle de l'action du Gouvernement. Dans le système actuel, nous passons effectivement trop de temps à discuter des effets anticipés d'une disposition, et trop peu à les vérifier. Nous adorons prédire le meilleur ou le pire pour une réforme, mais rechignons souvent à quantifier et à qualifier ses échecs ou ses succès. Il n'est pas sain, pour notre démocratie, de sembler n'avoir pas de suite dans les idées. Il n'est pas sain que le Gouvernement n'ait pas plus à rendre compte de son action auprès de la représentation nationale. Il n'est pas sain, donc, que le Parlement ne marche que sur une jambe. La représentation nationale doit pouvoir mieux assumer le deuxième versant de sa mission constitutionnelle : le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Je sais le Sénat très désireux d'améliorer la capacité du Parlement à suivre l'application des lois, à les évaluer dans la durée, à exercer sa mission de contrôle. Les discussions entamées cette semaine par le Premier ministre en vue de la révision constitutionnelle permettront précisément d'atteindre cet objectif et de renforcer cette évaluation. Je pense, par exemple, au rôle nouveau que pourrait assumer la Cour des comptes dans les missions d'évaluation et de contrôle du Parlement, ou encore à la possibilité d'enrichir la semaine de contrôle, d'en faire l'outil qu'elle aurait dû être depuis sa mise en place, au service d'un contrôle efficace de l'action du Gouvernement et du suivi de l'application des lois. Je l'ai dit lors de ma précédente intervention : nous devons rééquilibrer le travail et le calendrier parlementaires, favoriser notamment la tenue d'un débat budgétaire de printemps consistant, efficace, permettant de suivre l'application des lois dans la durée et d'analyser au mieux les résultats de l'action gouvernementale.

La présente proposition de loi tend à créer une délégation parlementaire dénommée « conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être », sur le modèle de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, l'OPEL, et de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, l'OPEPP, communs aux deux assemblées et tous deux créés en 1996. L'OPEPP a été supprimé en 2000, l'OPEL en 2009. Ce dernier a produit, en tout et pour tout, trois rapports en treize ans, malgré des moyens importants. Cela laisse à penser que la formule retenue n'est peut-être pas la bonne.

Il semble surtout que l'option déjà retenue par le Sénat de confier aux commissions permanentes le soin de veiller au suivi et à l'évaluation des lois soit plus pertinente et plus efficace. En effet, c'est en leur sein que se trouvent déjà toutes les compétences nécessaires à un suivi efficace des textes adoptés. Il est parfaitement logique de confier à la commission qui a longuement travaillé à l'élaboration d'un rapport, qui a ensuite voté un texte, qui s'est positionnée sur des amendements, le soin de se pencher ensuite, plusieurs mois ou années après, sur l'application et l'évaluation

puisse en suivre l'application pendant toute la durée de son mandat. Je ne peux m'empêcher, monsieur le rapporteur, en écho à votre intervention, de souligner que le secrétariat général du Gouvernement est désormais chargé

Si le Gouvernement a des propositions fortes à faire au Parlement pour renforcer ses missions de contrôle et d'évaluation, il compte aussi sur le Parlement pour se saisir de ses pouvoirs et trouver les meilleures solutions pour renforcer son action de contrôle et d'évaluation. La seconde question posée par cette proposition de loi a trait aux critères retenus pour mener à bien une évaluation satisfaisante des politiques publiques. S'il ne revient pas au Gouvernement d'interférer dans le choix des méthodes retenues par le Parlement pour évaluer les lois et les politiques publiques, je puis du moins vous assurer, mesdames, messieurs les sénateurs, que les nouveaux indicateurs de richesse prévus par la loi dite « Sas », que la présente proposition de loi veut promouvoir, sont d'ores et déjà largement pris en compte dans de nombreuses administrations. Ainsi, à Bercy, les indicateurs de niveau mission, qui rendent compte des grandes priorités des politiques publiques conduites par le Gouvernement, sont, pour la plupart, mis en cohérence avec ces nouveaux indicateurs de richesse dans les projets annuels de performance depuis 2017. Dans la troisième édition du rapport annuel sur les nouveaux indicateurs de richesse, publiée voilà deux semaines, le Gouvernement s'est engagé à aller encore plus loin. Comme l'a annoncé le Premier ministre, « dès l'année prochaine, les principales réformes engagées par le Gouvernement seront ainsi évaluées à l'aune de ces indicateurs pour juger de leur adéquation avec notre volonté d'engager la France vers une croissance plus verte et plus inclusive ». L'Assemblée nationale et le Sénat ont également pris les choses en main, avec la mise en place, au sein de leurs commissions du développement durable respectives, d'un groupe de travail chargé d'examiner les expériences étrangères de présentation du budget à l'aune d'objectifs de développement durable. Nous ne sommes encore qu'au début de l'aventure, mais les chantiers sont lancés, et l'ambition politique est là. Nous constatons qu'elle est partagée. Vous l'aurez compris, le Gouvernement estime utile la contribution de cette proposition de loi au débat sur l'évaluation des politiques publiques. Il est tout à fait vertueux que, dans cette période particulière de la législature- la première année, si importante pour les relations entre le Gouvernement et le Parlement, dans un moment essentiel pour l'avenir de nos institutions, celui des consultations menées par le Premier ministre en vue de la révision constitutionnelle -, nous prenions le temps du dialogue, de l'échange de vues sur des points qui structureront notre travail en commun. C'est ainsi que, avec la commission des lois et son rapporteur, nous considérons cette proposition de loi comme un texte utile au dialogue et à la réflexion, mais probablement insuffisant pour répondre pleinement à tous les enjeux de l'évaluation des lois. C'est la raison principale pour laquelle le Gouvernement soutiendra la motion de la commission des lois tendant au renvoi du texte à la commission.

le bien-être présent dépend à la fois des ressources économiques comme les revenus et des caractéristiques non économiques de la vie des gens : ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire, leur appréciation de leur vie, leur environnement naturel le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, établi en 2008, définissait le « bien-être présent », qu'il distinguait de la soutenabilité. Depuis la publication de ce rapport commandé par le président Sarkozy et destiné à améliorer la mesure des performances économiques et du progrès social, peu d'initiatives législatives ont visé explicitement à mettre en oeuvre ses recommandations. Elles s'adressaient en effet en premier lieu aux instituts produisant les statistiques à partir desquelles sont construites nos politiques publiques, ainsi qu'à la communauté scientifique, afin que soit mieux prise en compte la pluridimensionnalité du bien-être. Il est important de le souligner, les auteurs du rapport, tous d'éminents membres de la communauté des chercheurs, avaient conscience d'ouvrir un long débat, destiné à « aborder les valeurs sociétales auxquelles nous attachons du prix et déterminer dans quelle mesure nous agissons réellement en faveur de ce qui importe Ces préconisations continuent donc de faire leur chemin : le Parlement s'est récemment saisi de la question, en adoptant la loi du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

La valeur absolue de l'indice calculé par le PNUD s'est également affaiblie, passant de 0,93 à 0,89. C'est à juste titre que les auteurs de cette proposition de loi cherchent à prolonger le débat ouvert en 2008, même si les évolutions suggérées ne nous paraissent pas totalement satisfaisantes. d'abord, le rapporteur a rappelé l'échec des précédents organes parlementaires dédiés à l'évaluation des politiques publiques, avec les suppressions successives de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques et de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, en 2000 et en 2009. La création d'un conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être, à la composition certes innovante, semble viser à ressusciter ces offices, sans que rien permette de penser qu'il ne subirait pas le même sort.

et à permettre la production de contre-expertises au rapport publié au moment de l'examen de la loi de finances, en application de la loi de 2015 déjà citée. Ces dispositions ont le mérite de souligner que la prise en compte d'autres indicateurs que le PIB doit être constamment recherchée, tout au long de la chaîne d'élaboration de nos politiques publiques. Elles passent cependant à côté du problème central, à savoir le déficit d'intégration de critères qualitatifs de croissance lors des arbitrages politiques et budgétaires.

Certains se sont par exemple étonnés que, en 2017, l'indice de développement humain de la Libye, alors en guerre, tel que calculé par le PNUD, ait été supérieur à celui du Maroc Afin d'accroître l'influence des nouveaux indicateurs de bien-être proposés dans le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, il aurait été intéressant de les intégrer à la liste des éléments devant figurer dans les études d'impact prévue à l'article 8 de la loi du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Une autre piste à explorer serait le renforcement des liens entre le monde universitaire et les personnes chargées d'élaborer les politiques publiques françaises et européennes. De nombreux chercheurs français se distinguent sur la scène scientifique internationale dans des domaines concernés par les recommandations de la commission Stiglitz, qu'il s'agisse de l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, de l'évaluation des inégalités, de la prise en compte des activités non marchandes ou encore de l'évaluation de la soutenabilité. Il serait utile de réfléchir à des mécanismes qui permettraient de mieux tenir compte de l'ensemble des résultats de leurs recherches, au-delà des analyses produites par les chercheurs d'instances telles que le Conseil d'analyse économique. Enfin, la présence de pays à faible densité de population comme la Norvège et le Canada en tête des classements mesurant le bien-être me conduit à penser que cette dimension devrait également être mieux prise en compte en France, dans le cadre de notre politique d'aménagement du territoire. Trop souvent, le mal-être lié aux grandes concentrations de population est sous-estimé dans nos politiques publiques. Malgré tout l'intérêt du sujet abordé au travers de cette proposition de loi,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2008, le gouvernement français sollicitait la création de la Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social, dans un contexte de remise en cause croissante de la pertinence des indicateurs de performance économique et de progrès social existants. Cette commission, présidée par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, était chargée de déterminer les limites de l'utilisation du PIB comme indicateur de performance économique et de progrès social. De fait, il s'agissait d'une critique formelle de l'utilisation du PIB en tant qu'instrument de mesure central de la « richesse des nations ». Ainsi, dans son rapport final, la commission concluait que « l'adéquation des instruments actuels de mesure des performances économiques, notamment de ceux qui reposent uniquement sur le PIB, pose problème depuis longtemps ».

», a été l'occasion pour l'ONU de proposer un indice de richesse globale, « PIB vert » intégrant un « capital naturel » au PIB classique.

Cette loi prévoyait la prise en compte de dix nouveaux indicateurs de qualité de vie et de développement durable pour l'élaboration des décisions publiques, en sus d'instruments de mesure de la production tels que le Dans cette optique, elle impose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport annuel présentant l'évolution, à moyen terme, de ces indicateurs de qualité de vie et de développement durable. C'est dans la continuité de ces différentes initiatives que s'inscrit la proposition de loi de notre collègue Franck Montaugé.

Cette délégation parlementaire serait appuyée par un comité scientifique composé d'universitaires et de représentants d'organismes publics et indépendants. Elle devrait organiser de façon annuelle une conférence «

et du bien-être présente tous les trois ans un rapport- un de plus ! - évaluant la pertinence des indicateurs de richesse existants et formulant des propositions d'amélioration de ces derniers et de création de nouveaux indicateurs « plus qualitatifs ». l'article 3 dispose que le rapport gouvernemental visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques prévu par la loi devra désormais inclure une contre-expertise réalisée par des experts indépendants.

ouvre une réflexion intéressante sur la pertinence du PIB. Toutefois, mes chers collègues, gardons à l'esprit que la multiplication de structures en tout genre ne saurait constituer à elle seule une solution satisfaisante.

l'utilisation des nouveaux indicateurs à des fins d'action publique ou de pilotage des politiques publiques se révèle encore limitée. Enfin, les auteurs de la proposition de loi préconisent que le rapport gouvernemental présentant

de loi prévoit la création d'un conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être chargé d'« informer le Parlement sur la politique suivie [ ...] au regard des nouveaux indicateurs de richesse

non seulement d'informer le Parlement des conséquences des politiques publiques sur le bien-être des populations, mais aussi de mettre en place une plateforme participative numérique relative aux « nouveaux indicateurs de richesse afin que les citoyens s'approprient les indicateurs alternatifs au PIB et fassent vivre le débat démocratique. Cette plateforme a pour vocation l'élaboration et la mise en débat citoyen les nouveaux indicateurs, afin de rétablir le lien entre politiques et citoyens et d'attirer l'attention, notamment des médias, sur l'état de la société au travers des grands enjeux démocratiques. À cet effet, le conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être organiserait chaque année au Sénat une conférence citoyenne sur l'état des inégalités en France. L'article 2 de la proposition de loi instaure un bilan d'évaluation de la pertinence des nouveaux indicateurs de richesse

Ainsi, tous les trois ans, le conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être évaluerait la pertinence des indicateurs de richesse existants. Il formulerait des propositions d'amélioration ou de création de nouveaux indicateurs. Enfin, l'article 3 de la proposition de loi prévoit que le rapport issu de la loi Sas et remis par le Gouvernement au Parlement fasse l'objet d'une contre-expertise indépendante. Plus simple, il n'y a pas ! Cette proposition de loi appelle un certain nombre de remarques. En premier lieu, l'évaluation et le contrôle sont au coeur de la mission du Parlement, comme le dispose l'article 24 de la Constitution. Cette fonction vise à garantir la qualité des textes de loi en amont

afin d'améliorer l'évaluation de l'application des lois et, plus largement, l'évaluation des politiques publiques. Cette mission appartient aux commissions permanentes, ainsi qu'aux délégations et autres organes permanents ou temporaires. En second lieu, de nombreuses réflexions sur le renforcement du contrôle et de l'évaluation ont été entreprises et, déjà, des pistes ont été dégagées. Ainsi, il paraîtrait intéressant de renforcer l'assistance de la Cour des comptes. Actuellement, seules deux procédures permettent aux instances parlementaires d'être à l'initiative et de passer commande à la Cour des comptes d'enquêtes sur des sujets de leur choix. Il s'agit, d'abord, de la faculté reconnue aux commissions des finances, puis aux commissions des affaires sociales, d'user d'un droit de tirage dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit, ensuite, de la possibilité ouverte au président de chaque assemblée de demander la réalisation d'enquêtes au titre de l'évaluation des politiques publiques. Étendre à toutes les commissions permanentes la faculté de solliciter la Cour des comptes pour la réalisation d'enquêtes peut constituer une piste intéressante. De même, lever l'interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d'enquête sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires, sous réserve du respect du secret de l'instruction, peut sembler pertinent. La création d'une commission d'enquête est un outil essentiel du contrôle parlementaire. Toutefois, une règle de recevabilité prohibe la création d'une commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle était chargée d'enquêter. Le respect de cette règle repose, dès lors que la création d'une commission d'enquête est envisagée, sur une saisine systématique du garde des sceaux. Cette règle de recevabilité a, par le passé, limité les investigations des commissions d'enquête consacrées au Service d'action civique, aux sectes, au régime étudiant de la sécurité sociale ou encore au Crédit lyonnais,

Enfin, prévoir un délai impératif de réponse de deux mois aux questions écrites posées par les parlementaires au Gouvernement irait dans le sens d'une valorisation des activités de contrôle et d'évaluation du Parlement. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ces quelques exemples illustrent des voies d'amélioration et de développement des travaux d'évaluation. Dans ce contexte, la proposition de loi visant à instituer un conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être apporte une contribution utile.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'indicateur du PIB a été instauré en 1945, aux fins de quantifier les besoins des Français, en pleine période de reconstruction. Il s'agissait alors de mesurer le développement de la société, ses progrès, avec l'objectif presque exclusif d'apprécier sa capacité à produire toujours plus de richesses. Cet indicateur, aujourd'hui au service de la compétitivité, vieux de plus de soixante-dix ans, a besoin d'évoluer en profondeur. En effet, le PIB souffre de plusieurs lacunes : il ne mesure pas la répartition des richesses dans la société ; il ne prend pas en compte les ressources naturelles des pays, en termes énergétiques ou de biodiversité

de sa population, être à l'écoute des citoyens et cesser de se focaliser uniquement sur les enjeux économiques, comme cela a pu être le cas par le passé. Ce constat est aujourd'hui largement partagé, sur tous les bords politiques. Nicolas Sarkozy, en 2008, avait installé la commission Stiglitz, dite « commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social ». Cette commission avait engagé une réflexion sur les moyens d'échapper à une approche trop quantitative, trop comptable, de la mesure de nos performances collectives.

la prise en compte de dix nouveaux indicateurs de richesse, qui donnent lieu à la publication d'un rapport annuel permettant d'évaluer l'état de la France. Plus récemment, le député du « nouveau monde » Bruno Bonnell- j'ai parcouru l'ensemble du spectre politique ! -s'est créé une certaine notoriété en déclarant On n'entend que ça, le pouvoir d'achat, comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter ». Même si je suis en désaccord total avec M. Bonnell en ce qui concerne sa conclusion, je crois, comme lui, comme M. Sarkozy, comme Mme Sas et comme M. Stiglitz, que nous aurions beaucoup à gagner à utiliser des indicateurs plus adaptés à nos évolutions sociétales. Quels sont les indicateurs à retenir ? Quelles seraient les conclusions que nous pourrions tirer des nouvelles tendances ? Nous n'en savons encore rien. Une telle évolution permettrait-elle de dissimuler la question du pouvoir d'achat, comme le souhaite M. Bonnell ? Permettrait-elle de mettre au jour de nouvelles inégalités, comme l'estime Amartya Sen, qui déclarait en 2009 : « Les indicateurs de production ou de consommation de marchandises ne disent pas grand-chose de la liberté et du bien-être, qui dépendent de l'organisation de la société, de la distribution des revenus. La loi Sas avait défini dix nouveaux indicateurs. Actuellement, nous ne pouvons pas, avec le seul indicateur qu'est le PIB, anticiper l'impact d'une décision sur l'écologie

Le PIB mesure le niveau de vie du pays ; c'est donc un indicateur qui évalue, mais qui ne porte pas d'ambition sociale ou transformatrice. Les dix indicateurs de la loi Sas étaient le taux d'emploi, l'effort de recherche, l'endettement, l'espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie, les inégalités de revenus, la pauvreté en conditions de vie, les sorties précoces du système scolaire, l'empreinte carbone, l'artificialisation des sols. ces indicateurs vise donc à changer les pratiques du Gouvernement, à le forcer à prendre en compte des indicateurs qu'il négligeait, afin de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Selon les mots d'Édouard Philippe- vous voyez, mes chers collègues, que j'ai toujours de bonnes références -dans le dernier rapport sur ces indicateurs de richesse, Cette dynamique n'est pas un travail en chambre, elle n'est pas simplement un exercice de spécialistes, elle a un sens politique profond. Il s'agit de savoir ce sur quoi nous fondons collectivement notre appréciation de ce que nous entendons par les termes de croissance, de développement, de bien-être ou de progrès Il est vrai que certains de ces indicateurs sont plus difficilement mesurables, comme le niveau de satisfaction dans la vie. Bien que les réponses apportées soient subjectives, elles n'en restent pas moins révélatrices de l'état actuel de notre société ; à ce titre, les valeurs en question sont à prendre au sérieux. Il y a donc les indicateurs, et ces nouveaux indicateurs sont une très bonne avancée. Il y a aussi, et c'est tout aussi important, notre capacité collective à les évaluer : non pas comme le fait le Gouvernement, c'est-à-dire de manière annuelle, en mesurant les résultats établis durant l'année, mais dans leur efficacité, leur utilité, leur impact concret. Nous pensons qu'il est important de faire un bilan d'évaluation sur la pertinence de ces indicateurs, avec la possibilité de les compléter, donc d'en ajouter, afin de les rendre plus complets et plus exhaustifs. Pour vous donner un exemple, nous pourrions ajouter aux indicateurs existants des « blocs d'indicateurs ». Serait ainsi créé un indicateur de soutenabilité sociale, qui regrouperait des indicateurs d'inégalités fondés sur des indicateurs de répartition, mesurant les inégalités de revenus, les inégalités territoriales- elles ont été citées tout à l'heure -concernant l'accès aux dispositifs de l'État et les inégalités des chances. À ce premier bloc s'ajouterait la création d'un indicateur de l'état du patrimoine national, mesurant, donc, le capital productif de la France, son capital humain, son capital social, mais également son capital naturel, autant de mesures essentielles pour améliorer notre bien-être dans le futur. Enfin, un dernier bloc consisterait en un indicateur de responsabilité écologique de la France dans le monde, nous permettant de mesurer l'impact écologique de notre pays en recourant aux indicateurs d'empreinte carbone et de consommation carbone. Pour le moment, le rapport annuel présente l'évaluation de l'impact des principales réformes engagées par le Gouvernement, mais il est principalement utilisé dans le cadre des lois de finances. Un élargissement de son utilisation,

au moyen des indicateurs nouvellement adoptés. Afin de rendre ces indicateurs vraiment efficaces, une évaluation plus qualitative des projets de loi, l'intégration des nouveaux indicateurs de richesse dans les Un renforcement de la prise en compte des nouveaux indicateurs mettrait en lumière ces derniers et permettrait de mieux prévoir les incidences des lois futures sur la vie de nos concitoyens. Nous proposons Nous proposons en outre, le texte de Franck Montaugé, que le rapport annuel issu de la loi Sas, qui est remis par le Gouvernement au Parlement, puisse faire l'objet d'une contre-expertise indépendante. Cette proposition est importante. En effet, le rapport est actuellement rédigé par les services du Premier ministre et vise à évaluer la politique du Gouvernement, ce qui peut créer des conflits d'intérêts et conduire à négliger certaines données révélées par les indicateurs.

Permettre au Parlement de demander une contre-expertise irait dans le même sens, celui du contrôle accru des actions du Gouvernement, et octroierait plus de légitimité aux résultats dudit rapport, la proposition de création d'un Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être de notre collègue Franck Montaugé. Composé de dix-huit députés et de dix-huit sénateurs, ce conseil aurait pour ambition de tenir le Parlement informé des conséquences des politiques publiques sur le bien-être des populations,

service public, la qualité de l'air, etc., avec des données plus précises. Elle serait beaucoup plus importante que de simples rapports annuels, dont nous mentirions, mes chers collègues, si nous affirmions que nous les dévorons tous ...

L'évaluation des politiques, angle mort de notre vie publique, nécessite de la créativité. Dans cette perspective, avec sa proposition, Franck Montaugé fait oeuvre utile. utile. Il manifeste, avec ses deux textes, une impatience qui fait honneur au Parlement et qui vient répondre à une demande sans cesse formulée : c'est souvent « pour demain », ce n'est jamais le moment ... Aujourd'hui, c'est la question de la réforme constitutionnelle qui nous amène à différer ce travail.

que nous propose Franck Montaugé. Nous ne nous opposerons pas au renvoi en commission, pleins d'espoir dans le travail à venir, mais nous nous abstiendrons avec sagesse, en attendant que soient enfin pris ces indicateurs de richesse et engagées ces politiques d'évaluation que l'on nous promet toujours et qui n'arrivent jamais. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, on ne peut évidemment s'en remettre à la seule création de richesse pour mesurer la bonne santé d'un pays et de ses habitants il est absolument nécessaire de s'assurer de la pérennité et des impacts des politiques publiques en procédant à leur évaluation. Ces politiques doivent répondre à un objectif de développement durable, ou soutenable, tel qu'il a été défini en 1987 par la Commission mondiale pour l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies : « [ ...] Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs Lorsque l'on s'intéresse à un pays, la focalisation sur la seule création de richesses ne reflète absolument pas la réalité du niveau de vie de ses habitants. À l'idée fausse qu'une performance économique entraîne nécessairement une amélioration des conditions sociales, il manque, entre autres, une information sur la répartition de la richesse créée, en écart de rémunération et de patrimoine bien sûr, mais surtout en termes de possibilité pour chacun d'accroître sa Le critère pécuniaire n'est toutefois pas le seul à prendre en compte dans l'estimation de la qualité de vie d'un individu. Il faut en effet s'intéresser aussi aux facteurs physiques, psychologiques et sociaux, éléments constitutifs du bien-être d'une personne l'espérance de vie en bonne santé, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les liens sociaux, l'accès à l'éducation pour ses enfants, ou encore le respect des droits fondamentaux. L'idée d'ajouter une telle grille de lecture au calcul de la richesse d'un pays et à l'évaluation des politiques publiques est tout à fait pertinente. Il est essentiel également d'inclure dans l'analyse des évaluations de soutenabilité des politiques économiques, afin d'avoir une vision plus prudente de leurs résultats. ainsi de prévenir de nouvelles crises, comme celle qui est survenue en 2008, lorsque les performances en apparence brillantes de l'économie mondiale entre 2004 et 2007 se révélèrent avoir été obtenues au détriment de la croissance à venir. En ce sens, la présente proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être, présentée par notre collègue Franck Montaugé, va dans le bon sens : elle tente d'apporter une réponse à ces différentes préoccupations. Le dispositif proposé, néanmoins, n'est pas satisfaisant.

créés en 1996 et supprimés depuis lors, après n'avoir publié que très peu de rapports et avoir souffert des discordances entre les majorités respectives des deux chambres. figure également la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, créée en 2011 et supprimée à son tour par manque de productivité. Créer encore une nouvelle structure exigera nécessairement un investissement supplémentaire de temps et d'énergie de la part des parlementaires. À force de dispersion, les élus finissent par travailler de manière moins efficace. Rappelons aussi que la mission d'évaluation des lois et des politiques publiques est normalement la prérogative des commissions permanentes. C'est très vrai ! C'est la raison pour laquelle l'OPEPS, avait été supprimé lui aussi, malgré sa production relativement importante, au motif que ses travaux pouvaient être menés au sein des commissions des affaires sociales de chaque assemblée.

aux arguments que j'ai invoqués lors de la présentation de mon rapport pour défendre cette motion de renvoi en commission. Cette motion est non pas une clause de style- j'ai fourni

à partir du point de départ que représente cette proposition de loi, sur cette question de l'évaluation des politiques publiques, et principalement de l'application des lois. Je pense, mes chers collègues, en avoir assez dit ! Personne ne demande la parole contre la motion

que le groupe de travail présidé par Gérard Larcher et dont François Pillet est le rapporteur, qui poursuit qui poursuit sa tâche pour déterminer les propositions du Sénat en matière de révision des institutions, a été parfaitement conscient du problème soulevé par cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle il a lui-même formulé des propositions que je crois extrêmement utiles, tant sur le renforcement des études d'impact, dont la substance n'a pas été suffisamment vérifiée par le Conseil constitutionnel et qui, de ce fait, est resté largement lettre morte, que sur l'évaluation de la mise en oeuvre des lois, notamment des dispositions réglementaires nécessaires. Notre assemblée, quand bien même elle adopterait cette motion, est donc déjà force de proposition. Elle pourra d'ailleurs traduire elle-même ses propositions dans les textes dont elle aura à discuter, améliorer la qualité de la loi par des études d'impact, pour renforcer l'indépendance du Parlement par rapport aux organismes gouvernementaux l'évaluation des effets des projets de loi adoptés et pour faire en sorte que l'abstention du Gouvernement dans la mise en oeuvre des lois par des décrets soit sanctionnée, notamment par les recours devant par les recours devant le Conseil d'État, sous astreinte, que pourront faire, au nom de leur assemblée respective, les présidents de chacune des deux chambres. Il est très important de le rappeler. Notre débat, en effet, s'inscrit dans un contexte qui est celui de la réforme et de la modernisation de nos institutions. Quand on parle de modernisation des institutions, le Sénat répond évidemment présent

dans la discussion générale de la qualité de leurs propositions et réitérer le souhait du Gouvernement de travailler plus avant sur la question de l'évaluation et de l'application. J'ai dit tout à l'heure que le Gouvernement